La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la mission d'information sur le thème : « Uberisation de la société : quel impact des plateformes numériques sur les métiers et l'emploi ? » Conformément à l'article 8 du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques ont été publiées. Elles seront ratifiées s'il n'y a pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

est ainsi libellé : La parole est à M. Henri Cabanel. Les forêts primaires et les forêts matures jouent un rôle crucial dans le stockage du carbone et abritent la biodiversité la plus dense, avec des milliers d'espèces, souvent rares ou menacées. Elles sont, de surcroît, plus résistantes aux aléas climatiques que les forêts secondaires. Or nous constatons une régression préoccupante des forêts primaires et matures. S'il n'existe plus de forêt primaire en métropole, la Guyane dispose de la plus vaste forêt primaire de France et de l'Union européenne, s'étendant sur 80 000 La protection de ces forêts constitue une priorité identifiée dans le cadre de la stratégie européenne pour la biodiversité, notamment en raison de leur rôle de puits majeur de carbone. Il est prévu de définir, cartographier, surveiller et protéger strictement les forêts primaires et anciennes encore présentes dans l'Union européenne. Le présent amendement vise à inscrire les forêts primaires et matures parmi les ressources forestières reconnues d'intérêt général.

et pas seulement dans les forêts primaires ou matures. Les jeunes forêts, par exemple, constituent un enjeu majeur de biodiversité pour les années à venir. Par ailleurs, cet amendement est partiellement satisfait, puisqu'il s'avère qu'une

la biodiversité quel que soit le type de forêt concerné. Existe, en outre, la stratégie pour les aires protégées, avec un renforcement de la protection des écosystèmes, notamment pour certaines forêts qui présentent un caractère subnaturel ou permettant l'expression complète du cycle forestier. J'ajoute, en clin d'oeil, la création prochaine de la réserve intégrale de près de 3 000 hectares au sein du parc national de forêts. Je souhaite appeler votre attention sur le fait que les termes « forêt primaire » et « forêt mature » ne font pas, à ce jour, l'objet d'une définition consensuelle et partagée.

renforcer la place de la forêt dans ce projet de loi. Par cet amendement, nous souhaitons hiérarchiser les objectifs de la politique forestière de l'État et de la gestion des propriétaires privés inscrits à l'article 19 D,

sur les 30 millions de plants plantés par an aujourd'hui, 20 millions sont des résineux. Ces essences d'arbres connues pour leur capacité à pousser très vite ont des effets nocifs sur l'écosystème des forêts. Alors qu'il est plus que nécessaire de reboiser avec des essences capables de s'adapter aux changements climatiques, les résineux ont une capacité d'absorption du dioxyde de carbone très faible, ce qui rend les forêts de plus en plus vulnérables. Ainsi, cet amendement, proposé parDéclic etGreenlobby,vise à intégrer dans le nouveau code forestier cette nécessité de reboiser nos forêts de manière variée, afin de les adapter au mieux aux bouleversements climatiques.

lequel passe par un mélange d'essences et, donc, par des résineux. Je rappelle que nous avons besoin de ces résineux pour atteindre l'objectif de la stratégie nationale bas-carbone en matière de construction et de matériaux bois.

du fait de la déforestation, des incendies de forêt et de l'élevage. Le groupe d'amitié France-Brésil, que j'ai l'honneur de présider, y est particulièrement sensible. L'urgence est donc non seulement climatique, mais, plus largement, environnementale, car climat et biodiversité sont étroitement liés. Cette urgence impose des actions fortes et rapides. Surtout, cette urgence est mondiale ; elle concerne tous les pays et tous les habitants de la planète. Chaque État est responsable ; dans ce contexte, la France peut et doit montrer l'exemple. Les générations futures s'en souviendront. Le présent amendement vise à inscrire, dans le code forestier, les objectifs de conservation et de renforcement du puits de carbone forestier, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de la France à l'horizon de 2050. En effet, comme le souligne l'association Canopée, l'engagement de la France pour tenir les objectifs de l'accord de Paris doit apparaître dans le code forestier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cet état de fait conduit à une lacune absolument considérable : cet engagement n'est pas suffisamment pris en compte dans la politique nationale forestière retranscrite dans le programme national de la forêt et du bois. Or, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone que nous nous sommes fixés, il est essentiel de renforcer le puits de carbone forestier, ce qui doit se traduire concrètement par un plafonnement du niveau de prélèvements. Tel est le sens de notre amendement. La parole

voire de renforcement du puits de carbone forestier, indispensable pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de la France à horizon de 2050. Cet engagement de la France au titre de l'accord de Paris n'apparaît pas, actuellement, dans le code forestier. Il n'est, de ce fait, pas pris en compte à la hauteur des enjeux dans la politique nationale forestière retranscrite dans le programme national de la forêt et du bois. Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, il est essentiel de préserver, voire de renforcer le puits de carbone forestier, ce qui doit se traduire concrètement par un plafonnement au niveau des prélèvements dans les objectifs de la politique nationale forestière retranscrite dans le programme dans le programme national de la forêt et du bois. Selon le rapport annuel 2019 du Haut Conseil pour le climat, pour la période 2015-2018, le puits net de carbone du secteur des terres a diminué de 2,1 % par an en moyenne, du fait des forêts. Pourtant, la trajectoire de la stratégie nationale bas-carbone anticipait un accroissement annuel de 11 %. Le rapport annuel 2020 indique que cette tendance se poursuit. Les études françaises récentes sur le bilan carbone des scénarios d'augmentation de la récolte confirment les résultats à l'échelle européenne : une augmentation massive de la récolte augmentera les émissions de CO2 pendant au moins trois décennies. leur côté, les climatologues estiment que seule une diminution totale, d'ici à 2030-2050, peut nous permettre de rester sous le seuil de 1,5 degré de réchauffement ciblé par les accords de Paris.

les prélèvements forestiers dégagent du carbone leur impact sur le sol et, lorsqu'il s'agit de bois énergie, leur combustion. Ces émissions ne sont compensées par la repousse des arbres et la restauration du sol que des dizaines, voire des centaines d'années plus tard. Or c'est maintenant, dans les décennies à venir, qu'il nous faut réduire notre impact carbone. Le plafonnement proposé par cet amendement est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques de la France. Il correspond, par ailleurs, aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Si une confusion est entretenue à ce sujet, permettez-moi de dire et non les forêts jeunes, qui stockent le plus de carbone, notamment du fait du stockage dans les sols forestiers. En forêt tempérée, les sols stockent plus de carbone que la partie aérienne de l'arbre. En France, 79 % des arbres ont moins de cent ans et, donc, sont jeunes. Accélérer les prélèvements ne fera qu'accentuer la perte de stockage de CO2 par les forêts. De plus, une augmentation des prélèvements dégraderait la fertilité et la biodiversité des écosystèmes forestiers, hypothéquant ainsi nos chances de restaurer un bon état écologique des forêts françaises.

des émissions françaises. Ce puits est principalement constitué des écosystèmes forestiers, qui, en plus de fournir le bois nécessaire à la transition bas-carbone, séquestrent près de 87 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 19 des émissions annuelles françaises. Le rôle de puits de carbone de la forêt a été inscrit par d'autres dispositions au sein de notre politique forestière nationale. Nous proposons,

J'ajoute que, en associant les effets du puits forestier et l'augmentation du stockage des produits bois, nous activons aussi ce troisième levier de la substitution, qui doit nous permettre de répondre aux matériaux plus énergivores et aux

Cet amendement vise à consacrer, dans le code forestier, la possibilité de laisser des surfaces forestières en libre évolution, lesquelles peuvent jouer un rôle intéressant dans notre stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. En effet, si l'exploitation économique des forêts a toute sa vocation pour la création de matériaux durables et d'énergie, elle empêche le plus souvent le vieillissement naturel des arbres. Or le stockage du carbone se réalise d'autant mieux

des forêts en libre évolution sont les supports de vie d'un quart de la biodiversité terrestre. La libre évolution permet aussi de garder des témoins du fonctionnement originel des forêts et constitue un laboratoire précieux d'observation pour la connaissance du fonctionnement des écosystèmes forestiers, notamment dans le cadre du changement climatique. Pour ces

Cette pratique se répand dans les forêts dites de « feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences et des âges d'arbre différents, et donc plus résilientes au changement climatique, malheureusement dans le seul but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux. Les forêts plantées après coupe rase sont moins résilientes face au dérèglement climatique, aux incendies ou encore à la prolifération d'insectes. Cet amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts qui ne font pas actuellement l'objet d'une définition au sein du code forestier. Elles seraient ainsi définies « comme les coupes d'un seul tenant de la totalité des arbres d'une parcelle sans régénération acquise, d'une surface supérieure à deux hectares ». Elles seraient interdites, sauf « autorisation délivrée par le représentant de l'État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière

1101. Cet amendement vise à interdire la coupe rase, qui consiste à abattre la totalité des arbres d'une parcelle d'une exploitation forestière. Aujourd'hui, la coupe rase, ou coupe à blanc, est une technique qui ne tient pas compte des limites et des fragilités du couvert forestier français et qui a des effets dévastateurs sur l'écosystème, les sols et les paysages. La coupe rase entraîne une perturbation anormale et brutale de l'écosystème forestier, accroît le risque d'une mauvaise régénération des essences- si précieuse -et la compaction et parfois l'érosion des sols, ce qui nuit à la bonne régénération naturelle et au bon ancrage des arbres plantés. Enfin, cette pratique forestière peut conduire à une modification profonde et brutale des mécanismes de ruissellement et du cycle de l'eau, ce qui se traduit par une pollution ou dégradation des cours d'eau, localement et en aval. La parole est à Mme

d'une surface supérieure à deux hectares, sauf autorisation du préfet de département et du CNPF. La pratique des coupes rases constitue un véritable préjudice pour le stock carbone carbone contenu dans les sols forestiers. Elle doit, à ce titre, être interdite. Une récente étude, publiée par la Commission européenne en juin 2020, a révélé que la surface de forêt recollée par coupe rase avait augmenté de 49 % sur la période 2016-2018

de la surface forestière française en 2016. Ces chiffres doivent nous alarmer sur la nécessité d'endiguer ce phénomène afin de préserver notre surface forestière, dont le rôle est essentiel dont le rôle est essentiel pour la régulation du CO2 au niveau atmosphérique. Les forêts, qui stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées, doivent donc être protégées des coupes rases. La

après une coupe rase sont moins résistantes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d'insectes. Certes, la coupe rase,

avec de l'argent public ! -des pratiques qui consistent à détruire entièrement une forêt diversifiée, en parfaite santé, par coupe rase, puis à la remplacer par une autre plantation, généralement monoculture de résineux. L'industrialisation de la forêt se poursuit donc à rebours des enjeux sociétaux, environnementaux et économiques liés à ces milieux si précieux.

dans la loi, dans le code forestier, la préservation et la qualité des sols. Ce sont autant d'outils à la disposition des préfets et des CRPF pour contrôler

régionaux. Le code forestier permet aux préfets d'adapter le seuil d'autorisation des coupes d'un seul tenant, dites coupes rases, à un département, mais il ne permet pas de l'adapter à l'échelle d'un parc naturel régional (PNR). Cette incapacité d'adaptation aux enjeux spécifiques de ces territoires, pourtant particuliers sur le plan écologique et paysager, ne permet pas de répondre de manière efficace aux dynamiques identifiées dans les chartes de parcs, comme cela a été souligné lors de leur récente

tend donc à permettre aux préfets de département de fixer, en lien avec les syndicats mixtes à l'échelle d'un PNR ou d'une partie de PNR, un seuil d'autorisation de coupe de bois et forêts, comme ils peuvent le faire aujourd'hui à l'échelle du département. Les parcs naturels régionaux disposent d'une charte qui permet de justifier les objectifs d'une telle mesure et de définir la zone sur laquelle elle doit être mise en oeuvre.

que M. Labbé, peut-être pas avec la même fougue, mais avec la même détermination. Les coupes rases de forêts peuvent avoir des impacts très négatifs sur l'environnement : paysage, sols, biodiversité, cycle du carbone, cycle de l'eau

beaucoup de nos concitoyens exprimaient leur émotion devant ces coupes rases. Ces risques sont encore plus élevés dans les zones de montagne, car l'impact paysager est plus fort qu'en plaine, avec un risque accru d'érosion des sols. Dans les aires censées être protégées que sont les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, on constate aujourd'hui un manque d'outils juridiques pour réguler ces coupes. Cet amendement vise donc à mieux réguler cette pratique, en particulier dans les zones de

elles se définissent par un abattage de la totalité des arbres ou d'une parcelle d'une forêt. Cette pratique est malheureusement croissante, car nos forêts françaises sont en voie d'industrialisation : plantations, monocultures, coupes rases Cette pratique est pourtant contraire aux principes écologiques définis dans la Charte de l'environnement et en préambule du code forestier : « Sont reconnus d'intérêt général [ ...] la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; [ ...] la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone

comme puits de carbone. C'est le sens de notre amendement, qui tend à encadrer les coupes rases dans les zones de montagne, dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux. Quel

notion déjà incluse dans l'article 19 D. Comme je l'ai déjà souligné, le mélange des essences est un levier essentiel de la résilience des forêts françaises, fortement impactées par le changement climatique et les diverses crises sanitaires. Les monocultures, plus plus sensibles au changement climatique, aux tempêtes, aux invasions d'insectes, ont montré leurs limites dans de nombreux cas. Si de nombreuses incertitudes demeurent toujours sur l'adaptation des forêts au changement climatique, les scientifiques et les acteurs de terrain s'accordent sur un point pour améliorer la résilience des forêts au risque climatique et leur adaptation à des variations écologiques locales difficilement prévisibles, le maintien d'une diversité maximale

pour assurer, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, le renouvellement des peuplements forestiers respectent une diversité d'essences, en privilégiant les essences locales. Les schémas régionaux de gestion sylvicoles pourront définir les modalités de mise en oeuvre de cette disposition pour préserver une certaine souplesse et une bonne prise en compte des spécificités locales. libellé : La parole est à Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise également à assurer le renouvellement des peuplements forestiers après une coupe rase. La feuille de route pour l'adaptation de la forêt au changement climatique est assez claire : si la forêt a bénéficié pendant plus d'un siècle de conditions favorables à son développement, le changement climatique et son cortège de phénomènes extrêmes affectent désormais sa vitalité. Pour assurer la vitalité et la résilience de la forêt, notamment son adaptation à des variations écologiques locales difficiles à prévoir,

que les mesures prises après une coupe rase pour assurer le renouvellement des peuplements forestiers respectent une diversité des essences, en privilégiant les essences locales, afin d'adapter les forêts au changement climatique. Les schémas régionaux de gestion sylvicole définiront les modalités de mise en oeuvre de cette disposition pour préserver une certaine souplesse et une bonne prise en compte des spécificités locales. Quel

le stockage du carbone. Ils rendent à nos concitoyens qui vivent dans de grandes agglomérations un nombre important de services écosystémiques- cycle de l'eau, biodiversité, paysages

de protection », statut qui permet de protéger durablement les boisements et forêts. Une forêt est éligible à ce statut protecteur lorsqu'est reconnu son rôle pour la préservation de la sécurité des riverains contre certains risques naturels ou pour la santé et la qualité de vie des habitants de zones urbanisées, ou encore lorsqu'elle abrite des écosystèmes particulièrement particulièrement sensibles. Cette reconnaissance permet de la protéger, de la gérer ou de la restaurer en garantissant ses propriétés protectrices. Dès 1979, une circulaire du ministre de l'agriculture aux préfets indique que les principaux massifs forestiers proches des grandes agglomérations ont vocation à être classés en forêt de protection. Ce même objectif est explicitement mentionné et de la forêt, sur la mise en oeuvre de la politique relative aux forêts périurbaines, qui précise que l'action des préfets doit viser, pour ces forêts, « le classement progressif en forêt de protection des massifs les plus exposés ». Depuis, les pouvoirs publics ont régulièrement continué d'affirmer que le statut de forêt de protection était le plus adapté aux forêts périurbaines et à la lutte contre les pressions d'artificialisation qu'elles subissent. Pourtant, les forêts périurbaines ne bénéficiant pas de ce statut sont encore trop nombreuses. Dès lors, ce principe de classement des forêts périurbaines en forêt de protection mérite d'être porté au niveau législatif

Il faut en effet rappeler qu'actuellement 17,5 % de la récolte de chêne français est exportée en Chine du fait du moindre coût de la main-d'oeuvre dans ce pays. À l'heure où nous nous accordons tous sur la nécessité de relocaliser nos productions comme l'ont fait d'autres pays comme l'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie, le présent amendement vise à mettre un terme à cette pratique afin notamment de garantir l'avenir des petites et moyennes scieries

qui, contrairement à la récolte directe de bois en forêt, ne diminue pas le puits de carbone forestier. Transformer les grumes en France, c'est donc conserver ces coproduits sur le territoire et contribuer, leur valorisation, à diminuer l'empreinte carbone de la France.

de valeur tout au long de la chaîne : TVA, cotisations, fiscalité locale. Le départ des grumes hors Union européenne, qui est actuellement massivement pratiqué, est donc pénalisant pour les industries hexagonales, notamment pour les petites et moyennes, qui mériteraient de se développer mais sont privées de matières premières à transformer.

restriction à l'exportation de bois vers des pays tiers. J'ajoute que, malheureusement- vous le savez -, cette interdiction n'empêcherait pas l'exportation extracommunautaire de grumes, puisque l'essentiel des exports transite déjà par de grands ports situés en Europe du Nord, et ce au détriment de notre activité portuaire.

vote. J'ai un regret et une incompréhension : l'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie sont des pays européens

il faut faire attention à la Chine comme rival systémique.

et des résultats effectifs qu'ils obtiennent grâce à leurs changements de pratiques, ces PSE sont en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire. L'accompagnement technique et financier des agences de l'eau est financé un budget de 150 millions d'euros engagé sur trois ans,

pour l'avenir des travaux que nous menons ici et pour l'avenir de la forêt française : je veux parler de l'Office national des forêts, gestionnaire unique de nos forêts publiques, qui joue un rôle essentiel dans la préservation et l'administration de ces espaces naturels. Chacun le sait, les missions de l'Office sont nombreuses, variées, diverses : elles vont de la protection des milieux naturels et de la biodiversité à l'accueil du public en passant par la prévention des risques naturels et le développement de la filière bois énergie.

des tensions et même des conflits internes, la rentabilité étant difficilement conciliable avec l'exercice de missions d'intérêt général et de service public. L'hypothèse d'une procédure de filialisation de certaines activités suscite actuellement de vives inquiétudes. Les organisations syndicales, ainsi que d'autres parties prenantes, y voient un risque de démantèlement, à terme, de l'établissement. l'ONF, comme l'ensemble des autres opérateurs de l'État, est chaque année mis en difficulté et davantage affaibli par la poursuite de la diminution draconienne de ses effectifs. Près de 40 % de ses effectifs ont ainsi disparu en vingt ans, générant un malaise notable chez de nombreux salariés. Pourtant, pour que la France soit en mesure d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe en matière de politique forestière, elle doit mobiliser les moyens humains et financiers adéquats. Pour que l'ONF soit en mesure d'accomplir l'ensemble de ses missions, qui vont croissant, il doit donc disposer de moyens renforcés.

Nous ne pouvons évidemment pas le faire dans le cadre de ce texte, mais nous considérons que c'est un sujet primordial. Nous demandons donc, par cet amendement d'appel, que soit remis au Parlement un rapport sur l'adéquation des moyens financiers et humains mobilisés par l'État avec les objectifs

il y a déjà eu de très nombreux rapports sur les moyens consacrés à la forêt et à l'ONF ces dernières années. Le diagnostic est désormais bien connu : le bois n'a jamais suffi à payer

du conseil d'administration du 2 juillet de l'ONF sera présenté le nouveau contrat d'objectifs et de performance.

du modèle de financement, qui est nécessaire. Vous me demandez de vous éclairer sur ce sujet. Je crois que nous avons déjà entre les mains beaucoup d'éléments. Votre demande de rapport sur l'adéquation des moyens financiers et humains

Leur activité doit en effet être compatible avec l'objectif d'une gestion durable de la ressource en bois, en particulier avec la préservation du puits de carbone forestier et l'optimisation du bilan carbone Ce n'est bien sûr pas le seul levier susceptible de répondre à la dynamique observée, mais ce dispositif permettra tout de même d'apporter une première solution, en particulier en allant dans le sens de la préservation de nos ressources. Je vous confirme que l'ensemble du Gouvernement est fortement mobilisé sur ce sujet. Nous aurons sans doute à affiner ce dispositif, en étroite concertation avec la profession, mais nous souhaitons d'ores et déjà fixer ce marqueur, en réponse à la problématique actuelle.

Cet article, introduit par un amendement parlementaire à l'Assemblée nationale, vise à établir une stratégie nationale pour l'adaptation des forêts au dérèglement climatique. Cette proposition est louable, mais une feuille de route pour pour l'adaptation des forêts au changement climatique a été établie en 2020. Par ailleurs, l'article 19 F prévoit d'adapter le programme national de la forêt et du bois 2016-2026. Dans un souci de clarification et de simplification, il vous est demandé de supprimer cet article pour mieux le fusionner dans l'article suivant.

madame la ministre, ces deux articles dans un souci de lisibilité. Le programme national de la forêt et du bois est le document-cadre de la politique forestière. Il a vraiment vocation à porter les grands enjeux, dont l'adaptation des forêts. J'émets donc un avis favorable.

La commission est très attachée à l'article 19 F, qui doit permettre de réviser l'ensemble des objectifs du PNFB. Ces objectifs ne sont effectivement plus tenables après les crises et les dépérissements massifs

qui consiste à adapter le PNFB aux nouvelles réalités de nos massifs forestiers. Nous avions d'ailleurs publié en avril dernier une tribune invitant le Gouvernement à adapter sans tarder le PNFB aux nouvelles réalités liées au changement climatique. Nous souhaitons donc vivement un vote conforme sur cet article. Le PNFB, comme je viens de le souligner, est avant tout une stratégie de mobilisation du bois pour répondre aux besoins sociétaux. Il prévoit pour cela une augmentation des prélèvements à hauteur de 12 millions de mètres cubes d'ici à 2026, sachant qu'aujourd'hui nous n'exploitons même pas l'accroissement annuel de la forêt, celles-ci continuant donc à s'étendre, souvent au détriment des terres agricoles. C'est donc une stratégie au service du développement soutenable prenant en compte les enjeux environnementaux, économiques et sociaux

mois. Le problème du PNFB, comme nous l'avons évoqué, est qu'il a été établi en 2016, à partir de données encore antérieures et qui n'incluaient donc pas les impacts du dérèglement climatique, lesquels ont accéléré depuis les années 2017-2018. Le manque d'eau, associé aux très fortes chaleurs qui brûlent la cime des arbres, a affaibli les peuplements. Parallèlement, le réchauffement a favorisé la prolifération d'insectes ravageurs, comme les scolytes pour les résineux, mais aussi différentes espèces de chenilles pour l'ensemble des feuillus. Au final, aujourd'hui, toutes les essences d'arbre sont plus ou moins menacées. Plus de 10 millions de mètres cubes d'épicéas et de sapins ont déjà été atteints depuis trois ans, et ce n'est malheureusement pas terminé.

durablement les prévisions de récolte pour les années à venir. Il est donc inconcevable de rester avec les mêmes trajectoires de prélèvements dans les PRFB et le PNFB,

de ce programme, qui aura lieu en 2022. Une telle adaptation est une démarche lourde, qui risque de ralentir et de complexifier le PNFB.

Cet amendement est déjà satisfait par l'amendement n° 1831. S'il était adopté, il ferait perdre toute sa portée à l'article 19 F, car il offrirait la possibilité au Gouvernement non pas de réviser le PNFB, mais seulement de réviser un certain nombre de plans d'action.

À la différence de l'Hexagone, les forêts ultramarines ne font pas l'objet d'un suivi régulier et planifié au sein de l'inventaire forestier national. M. Falcone, adjoint au directeur général de l'Office national des forêts, et environnemental) le 22 septembre 2020, reconnaissait que l'impact du changement climatique est peu documenté concernant les écosystèmes forestiers en outre-mer, car il n'y a pas d'inventaire forestier en outre-mer, faute de moyens suffisants. octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a rendu obligatoire la prise en compte des ressources forestières nationales dans l'inventaire, ainsi que les particularités des bois situés en outre-mer. Or cette obligation n'est pas effective dans les territoires ultramarins. Les forêts ultramarines doivent faire l'objet du même niveau de connaissance, d'inventaire et de protection que les forêts de l'Hexagone. Leur préservation passe d'abord par la description détaillée de l'ensemble des essences et de la biodiversité. C'est pourquoi la réalisation d'un inventaire forestier complet par l'Institut national de l'information géographique et forestière tout comme la mise en place d'un réseau de suivi des écosystèmes forestiers équivalent au réseau Renecofor existant en France hexagonale sont nécessaires. De ce fait, cet amendement à portée programmatique générale vise à rappeler les engagements pris par l'État à l'égard des forêts des territoires ultramarins.

Les modalités de réalisation de l'inventaire en termes de méthodes ou de fréquences qui sont appliquées en métropole ne sont pas adaptées aux particularités des forêts d'outre-mer. Des études au cas par cas, des modalités spécifiques en fonction des enjeux à suivre sont, en l'espèce, à privilégier, d'où mon avis défavorable. Madame Schillinger,

de M. Patient est complémentaire du précédent. Il vise à inscrire dans l'article du code forestier qui instaure l'inventaire forestier national que celui-ci doit concerner tous les bois et forêts de France, y compris ceux d'outre-mer, ce qui jusqu'à présent ne semble pas encore être le cas. Par exemple, il n'y a pas d'inventaire en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que nous ne connaissons pas précisément les surfaces forestières de ces territoires. La couverture forestière des territoires ultramarins est pour la plupart d'entre eux supérieure à celle de l'Hexagone. La forêt guyanaise, qui est le plus

négatif à long terme de l'éolien offshore sur l'environnement. La mise en oeuvre de cette énergie risque en effet de nuire aux écosystèmes, à la biodiversité, au fonctionnement physique des bassins maritimes et, par conséquent, à la pêche artisanale côtière. Cet amendement vise ainsi à obliger l'autorité administrative chargée d'autoriser l'installation, l'exploitation et l'aménagement d'installations éoliennes en mer à rejeter une demande d'installation dans le cas où les conditions visant à préserver les ressources biologiques ne sont pas réunies, et ce au titre de l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Quel

territoriale, est déjà satisfait par la combinaison des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l'environnement.

de prendre en compte « la préservation des écosystèmes aquatiques [ ...], la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ». C'est pourquoi soumettre à une évaluation environnementale ces projets limiterait ce développement de l'énergie éolienne offshore à l'atteinte des objectifs de décarbonation de notre économie, alors que l'implantation d'éoliennes terrestres

nécessaire de mieux connaître les ressources souterraines pour se préparer aux défis de la raréfaction de la ressource. On le voit en effet, les étés sont de plus en plus secs, y compris dans les départements

L'article 19 , introduit à l'Assemblée nationale et non modifié lors de son examen en commission au Sénat, vise à inscrire dans les Sdage et les SAGE, c'est-à-dire les documents de planification dans le domaine de l'eau, l'identification et la protection des masses d'eau souterraines qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement. Cela suppose un nouveau dispositif de zonage et de nouvelles réglementations dans un millefeuille juridique qui est, avouons-le, déjà très complexe et particulièrement indigeste. Le principe de la priorité de l'alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages usages est incontestable, et il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet,

n° 511 rectifié. S'il est important d'identifier et de préserver les masses d'eau souterraines, il est également primordial de ne pas pénaliser l'activité humaine, notamment celle de nos agriculteurs, dont les conditions de travail sont déjà très difficiles. Face à cet enjeu, cet article pose trois problématiques majeures. Premièrement, il suppose la mise en place de nouveaux dispositifs de zonage et de nouvelles réglementations dans un millefeuille juridique déjà très complexe. Deuxièmement, comme l'a dit Stéphane Demilly, le Président de la République a annoncé en avril dernier le lancement du Varenne agricole de l'eau Ne serait-il pas plus judicieux d'attendre que soient rendues ses conclusions avant de légiférer ? Troisièmement, les risques de contentieux à l'encontre des activités agricoles que peut impliquer cet article sont disproportionnés. Nos agriculteurs pourront-ils continuer à prélever de l'eau pour l'irrigation dans ces masses d'eau ?

du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu'il adopte. Enfin, nous devons nous assurer de ne pas pénaliser les activités en lien avec ces masses d'eau souterraines, dont certaines peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés.

Il est pertinent de se doter d'une connaissance plus fine et cartographiée dans les Sdage des masses d'eau souterraines, afin d'anticiper de manière rationnelle la baisse prévisible des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable. Les arrêtés « sécheresse » concernent chaque été un nombre croissant de départements

Je constate que vos interrogations ne portent pas sur l'objectif de cet article, qui vise la protection des ressources en eau potable pour les populations actuelles et futures. Cet objectif, aucun d'entre nous ne peut y être indifférent. Vous vous interrogez plutôt sur l'articulation de cette disposition avec les outils actuels de protection des captages. Vous questionnez donc le caractère opérationnel de cet article. Sur ce point, je peux vous rassurer : les dispositions de l'article visent l'identification des aquifères stratégiques pour l'alimentation en eau potable, en s'appuyant sur les comités de bassin, qui sont les parlements locaux de l'eau et sont chargés, notamment, de l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle des grands bassins. Certains Sdage, notamment celui du bassin Rhône-Méditerranée, appliquent d'ailleurs,, depuis des années les dispositions de cet article. L'objectif est d'identifier, à l'échelle de l'aquifère, c'est-à-dire de l'ensemble de la nappe, les enjeux permettant d'assurer leur protection pour le futur. Les plans d'action concernés

La rédaction de cette disposition a été améliorée en séance à l'Assemblée nationale pour permettre une meilleure articulation avec le cadre législatif existant. À ce stade, le Varenne de l'eau n'apportera rien de plus sur ce point particulier. En effet, j'y insiste, il s'agit d'acquérir une connaissance dont nous avons besoin. Je ne crois pas qu'il soit urgent d'attendre. Bien au contraire, il est urgent d'avoir cette connaissance le plus tôt possible. J'émets donc un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

doute parfaitement louable. À force de complexifier les choses, je crains que l'on ne décourage les acteurs locaux et qu'à la sortie on n'avance pas très vite.

Si l'objectif est de préserver ces ressources stratégiques, il est essentiel que des zones de protection puissent être instituées, d'autant que l'article précise que des mesures peuvent être prises afin d'accompagner l'adaptation des activités humaines

n° 668 rectifié. Le principe de la priorité de l'alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu'une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité humaine, en particulier celles liées à la production alimentaire, en lien avec ces masses d'eau souterraines et aquifères, dont certaines peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres. En l'état de la rédaction de l'article 19 , les risques de contentieux à l'encontre des activités, notamment agricoles, dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l'eau pour l'irrigation dans ces nappes ? L'apport d'intrants pour permettre la production agricole, et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France, sera-t-il soumis à des mesures généralisées d'interdiction et à des risques de recours juridiques ? Les activités d'élevage risquent-elles, à terme, de se voir condamner ? Aussi, il est proposé de préciser que les mesures visées à l'article 19 sur l'équilibre quantitatif des prélèvements des masses d'eau souterraines prennent notamment en compte les besoins des activités humaines, plus particulièrement les activités de production alimentaire essentielles à la souveraineté alimentaire

commission ? Ces deux amendements visent à ce que les mesures prises pour la préservation des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable satisfassent en priorité les besoins pour la consommation humaine et les activités de production alimentaire, c'est-à-dire les prélèvements pour l'irrigation. Il paraît nécessaire de maintenir une « super priorité » pour les besoins de la consommation humaine. Celle-ci repose aujourd'hui sur l'article L. 211-1 du code de l'environnement, lequel dispose : « La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile

Citons l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou encore les programmes d'action spécifiques à l'échelle de l'aire d'alimentation du captage pour lutter contre les pollutions diffuses.

qui ont accueilli des activités industrielles ou minières a recommandé d'inclure dans le code de l'environnement des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. Notre objectif est de sécuriser la remise en état des sites et d'améliorer la surveillance des sols. Notre ambition, je le répète, est de toujours mieux prévenir et gérer les pollutions, ainsi que les risques sanitaires qui y sont associés. Nous avons traduit cette préconisation dans l'article 12 de la proposition de loi évoquée. De quoi s'agit-il ? Dans ses réponses au questionnaire de la commission d'enquête, la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection a relevé qu'à sa connaissance aucun arrêté ministériel des prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration ne fixait de contrainte et, donc,, de points de contrôle relatifs au suivi de la pollution des sols et des eaux souterraines. Dans ces conditions, nous souhaitons inclure des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines dans les arrêtés ministériels et dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux ICPE soumises à autorisation environnementale ou à enregistrement, mais non soumises à des obligations de rapport de base ou de surveillance régulière des eaux souterraines.

de la commission ? La commission d'enquête du Sénat sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, qui était présidée par Laurent Lafon et dont présidée par Laurent Lafon et dont la rapportrice était Gisèle Jourda, a effectué un travail très important. Certaines propositions figurant dans le rapport de la commission d'enquête ont d'ailleurs été reprises par le Gouvernement dans le projet de loi que nous examinons. Je pense à l'article 20 relatif à l'arrêt des travaux miniers, que nous examinerons dans quelques minutes. Ces amendements correspondent à la proposition n° 18 du rapport de la commission d'enquête et partent du constat de l'extrême difficulté technique de mesurer l'état de la pollution des sols.

Madame la ministre,

amendements visent à imposer une surveillance décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour l'ensemble des installations classées. Conformément à la directive IED, relative aux émissions industrielles, le code de l'environnement prévoit déjà pour les sites relevant de cette directive une surveillance périodique des sols et des eaux souterraines, au moins une fois tous les dix ans tous les cinq ans pour les secondes. Pour les autres sites soumis à autorisation ne relevant pas de cette directive et ceux soumis à enregistrement et déclaration, une surveillance éventuellement plus contraignante peut déjà être imposée pour des activités à risques pour les sols ou les eaux souterraines, par des arrêtés ministériels de prescription générale. Par ailleurs, au regard du dossier de demande d'autorisation ou d'enregistrement et des risques associés, ou sur la base d'un constat réalisé lors d'une inspection, le préfet peut prescrire à l'exploitant une surveillance régulière des eaux souterraines par les arrêtés préfectoraux d'autorisation ou d'enregistrement, y compris lorsque les installations ne relèvent pas de la directive IED.

garantira une capacité de relance beaucoup plus importante. Notre troisième axe, c'est la réunion des conditions d'une gestion réactive et transparente des risques sanitaires ainsi qu'une meilleure répartition des préjudices écologiques. Ce faisant, nous articulons

Joël Bigot, pour présenter l'amendement n° 1733 rectifié. Mieux prévenir et mieux gérer les pollutions des sols et les risques sanitaires qui y sont associés est une priorité : c'est l'une des ambitions de la proposition de loi visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France. vous êtes nombreux à avoir cosigné ce texte, et Mme Jourda vous en remercie. L'article 20 inscrit la prévention et la surveillance des risques d'atteinte à la biodiversité liés à la pollution des sols parmi les missions de l'Office français de la biodiversité. l'OFB assure notamment le développement de la connaissance, de la recherche et de l'expertise sur les espèces, les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre le changement climatique et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. Cet organisme nous semble le mieux placé pour remplir une mission de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines. Dans la continuité de ces travaux, nous voulons donc renforcer le rôle de l'OFB en matière de prévention et de surveillance des risques d'atteinte à la biodiversité en inscrivant au titre de ses missions le développement de la connaissance relative aux impacts de la pollution des sols sur la biodiversité. biodiversité. Ainsi, nous avons voulu traduire cette préconisation dans le présent texte. Malheureusement, l'article 40 nous en a empêchés. Nous voilà condamnés à demander un rapport sur les conditions d'élargissement des missions de l'Office français de la biodiversité. C'est bien dommage ! Madame la ministre, la connaissance de l'impact de la pollution et de l'artificialisation des sols sur les écosystèmes et la biodiversité mérite d'être approfondie. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir lors de ce débat, car l'artificialisation des sols fera partie des sujets que nous allons aborder.

de la commission ? Ces six amendements visent à demander la remise d'un rapport au Parlement sur les conditions d'élargissement des attributions de l'Office français de la biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines. Je ne suis pas favorable à un énième rapport : si la nécessité d'élargir les missions de l'OFB fait consensus, emparons-nous du projet de loi de finances pour confier aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'OFB la police de la qualité des sols et des eaux souterraines. J'émets un avis défavorable sur ces six amendements.

présenter l'amendement n° 304 rectifié. Avec cet amendement, nous proposons une expérimentation permettant aux collectivités territoriales de faire respecter la stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires d'autorisations d'urbanisme, en exigeant la preuve du bon respect des règles établies par le zonage pluvial. vise à permettre aux collectivités chargées de l'urbanisme, en coordination avec la collectivité chargée de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, de simplifier et de systématiser ces procédures au service de l'eau et de l'équité de traitement entre les porteurs de projet.

d'expérimenter diverses solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l'eau et de l'équité de traitement entre les porteurs de projet. Grâce

ces amendements proposent le lancement d'une expérimentation sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, portant sur la gestion des eaux pluviales à la source. Les autorisations d'urbanisme doivent d'ores et déjà respecter le zonage pluvial et les règles de gestion des eaux pluviales. Même si la vérification de leur respect ne fait pas l'objet d'une pièce spécifique dans le dossier de permis de construire, elles peuvent être contrôlées au titre des pièces existantes pouvant faire l'objet d'une demande de pièces complémentaires.

qui porte sur l'exploration et l'exploitation. Il a été significativement amélioré par l'Assemblée nationale, dont l'intention est plutôt bonne : il s'agit de rendre acceptables l'exploration et l'exploitation minières

du principe de précaution, du principe de réparation- ancien principe du pollueur-payeur -, du principe d'information et de participation ou encore de l'objectif de développement durable. Pourtant, en matière d'après-mine, les dégâts miniers et leurs victimes reconnus que très rarement, au terme de procédures judiciaires extrêmement longues et coûteuses. Même si le principe d'indépendance des législations ne peut plus être opposé à la pleine efficacité de la Charte constitutionnelle de l'environnement, il n'est pas inutile d'en rappeler la portée en précisant que les décisions prises dans le domaine du droit minier doivent tenir compte des principes structurant le droit de l'environnement. De nombreux territoires souffrent encore, des décennies après la fin de l'exploitation de leurs sous-sols. Pour tous les futurs bassins miniers, il est impératif d'avoir une meilleure gestion du risque environnemental qu'hier. Effondrements, pollution des nappes phréatiques, remontées toxiques, ennoyages et affaissements sont autant de conséquences observables de certaines exploitations minières.

à prendre compte tenu des données acquises de la science. L'objectif de développement durable doit être en filigrane de toute la réforme du code minier et du présent texte.

L. 161-1 du code minier, qui définit les intérêts protégés par ce code. Pour les carrières, l'article L. 511-1 du code de l'environnement permet d'assurer le respect des intérêts que vous visez. Aussi, rien n'impose d'introduire cette cette disposition dans le code minier. Par ailleurs, l'article 20 A, délégué au fond à la commission des affaires économiques, met en place un régime d'analyse environnementale, économique et sociale préalable à à l'octroi, à l'extension et à la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession. Ce régime permet également de satisfaire votre amendement : dès lors que le ministre ou le préfet, selon les cas, aura un doute sérieux sur la possibilité de procéder à la recherche ou à l'exploitation d'un gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés par le code minier, la demande de l'exploitant sera refusée. Je sollicite donc le retrait de ces amendements. À défaut,

argentifère. J'y avais travaillé, à l'époque, avec beaucoup d'associations et d'ONG, dont Ingénieurs sans frontières, mais aussi avec les peuples autochtones, notamment avec les Kali'nas de Guyane, qui mènent le combat contre la Montagne d'or, que vous venez d'évoquer,

quel impact ont les boues cyanurées à long terme, notamment dans la forêt amazonienne. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de projets de mines industrielles

très souvent recours à des produits dangereux à la fois pour notre santé, pour la biodiversité et pour l'environnement, et dont les conséquences sont souvent irréversibles. C'est le cas du cyanure, pourtant utilisé dans l'exploitation de minerais aurifères et argentifères. Son utilisation pour la lixiviation est mise en cause depuis de nombreuses années, notamment depuis la catastrophe de 2000 en Roumanie, qualifiée de pire désastre écologique en Europe depuis Tchernobyl. Ce déversement a contaminé l'eau potable de deux millions et demi d'Européens et a tué 100 tonnes de poissons et d'animaux sauvages, dont des espèces protégées. Il ne s'agit pas d'un accident isolé ; les cas de rupture de digues, de défauts de construction ou encore d'accidents de transport se sont multipliés ces dernières années. On en recense déjà vingt-cinq depuis 2000, soit plus d'un par an. Ces événements aux conséquences catastrophiques suffisent à justifier, aujourd'hui, l'interdiction de l'exploitation de minerais aurifères et argentifères

L'amendement que nous proposons ici répond non seulement aux ambitions de notre projet, mais également à celles de l'accord de Paris sur le climat ; de plus, il s'inscrit dans la continuité de la résolution du Parlement européen de 2017 demandant l'interdiction de l'usage du cyanure dans l'industrie minière en Europe. Certains pays européens l'ont déjà fait, comme l'Allemagne, qui a même anticipé cette résolution. Vingt ans après la fermeture de la mine de Salsigne, dans l'Aude, les habitants paient encore lourdement le prix de l'utilisation du cyanure, par l'industrie extractive. L'urgence environnementale implique de mettre un terme à l'utilisation de produits dont la toxicité n'est plus à prouver et de faire primer, par d'autres options, l'intérêt général de la santé humaine et de la préservation de notre planète. Quel

trois amendements. Ceux-ci portent sur l'interdiction du cyanure dans l'industrie minière, en particulier pour l'exploitation aurifère et argentifère. En France, cela concerne quasi exclusivement la Guyane. Le stockage et l'utilisation du cyanure présentent bien entendu des risques pour l'environnement,

des expérimentations -dont il serait scientifiquement démontré qu'elle a un meilleur impact environnemental que l'utilisation du cyanure. Des travaux sont menés sur le sujet- Mme la ministre pourra sans doute nous apporter des éléments complémentaires sur ce point -, mais, si nous adoptions ces amendements, nous ne pourrions pas continuer à mener des activités légales d'extraction d'or en Guyane de façon « convenable » ; je mets évidemment le rappelle, le projet de loi durcit la lutte contre l'orpaillage illégal et donc contre les techniques et les pratiques minières qui portent une atteinte forte à l'environnement et à la santé.

en effet entraîné des pollutions. Les normes appliquées aujourd'hui en France et en Europe sont les plus dures et les plus contraignantes concernant la conservation et l'utilisation du cyanure dans les mines.

de cyanure par an, mais aussi 6 600 tonnes de chaux, 100 tonnes de nitrate de plomb, 84 tonnes de soude, 1 800 tonnes de sodium, 60 tonnes de sulfates et 20 tonnes d'acide sulfurique. Or tout

des minerais d'or existent à l'échelle industrielle » ; « le procédé basé sur l'utilisation du thiosulfate atteint un niveau de maturité qui s'approche de la cyanuration. » Selon

Dans son rapport de 2017, le Parlement européen fournit une liste de douze technologies susceptibles de remplacer le cyanure, parmi lesquelles figure le thiosulfate, que nous venons d'évoquer, qui est utilisé à grande échelle par la

laquelle paraissait clairement insuffisante, et procède à un verdissement très attendu de ce code. Ont été insérés la préservation de la santé publique, la protection du littoral et du milieu marin ou encore les intérêts halieutiques. Le présent amendement vise à intégrer les intérêts forestiers à cette liste. Nous avons en particulier à l'esprit la Guyane, dont le territoire reste très convoité par les exploitants.

par ailleurs, la forêt guyanaise est également l'un des massifs forestiers français les plus importants, avec près de 8 millions d'hectares, et fait de la Guyane le département français le plus boisé. Selon le WWF, l'Amazonie européenne connaît, depuis plus de vingt ans, une nouvelle ruée vers l'or, dont les conséquences se révèlent désastreuses pour l'état forestier guyanais, malgré l'encadrement légal des exploitants déclarés. Il convient donc de renforcer la protection des forêts guyanaises contre les effets dommageables de l'activité minière française. Pour ce faire, cet amendement tend à compléter la liste des intérêts protégés requérant une demande d'autorisation d'ouverture des travaux en y intégrant les intérêts forestiers. Cette mesure paraît essentielle pour éviter que les forêts guyanaises ne subissent les attentes des exploitations minières déclarées, l'orpaillage illégal provoquant d'ores et déjà des dégâts colossaux sur l'environnement. de la commission ? Ces deux amendements me semblent satisfaits, dès lors que l'on considère que les intérêts agricoles couvrent également les intérêts sylvicoles, ce qui doit être le cas, à mon sens. Le fait de le dire expressément dans nos débats indiquera l'intention du législateur. La rédaction de l'article L. 161-1

Manque de bol, au bout de quinze ans, l'État, qui avait repris les installations, s'est rendu compte que les dispositifs adoptés étaient totalement insuffisants,

Cet amendement est satisfait, car l'administration procède à une contre-expertise de la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cette contre-expertise administrative permet ensuite au préfet de prescrire la réalisation de mesures à l'exploitant, puis de les contrôler lorsqu'il a donné acte de leur réalisation. Par ailleurs, il me paraît paradoxal et quelque peu problématique de faire financer cette contre-expertise par l'exploitant lui-même. Cela ne permet pas de garantir un respect du principe du contradictoire et de l'indépendance de notre administration

qu'un délai soit imposé pour la délivrance de l'arrêté de second donné acte à compter du procès-verbal de récolement et de réalisation des travaux.

amendement tend à revenir sur la prescription trentenaire. Lorsque les mesures d'après-mine ont été exécutées, l'autorité administrative en donne acte, ce qui met fin à l'exercice de la police des mines.

inférieure à la durée de validité du titre minier. Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer la prescription de trente ans, afin qu'il n'y ait plus de délai de prescription pour des dommages qui peuvent survenir plusieurs décennies après les travaux miniers ; nous avons tous des exemples en tête.

Ainsi, le territoire français compte plus de 3 500 anciennes mines, qui continuent, plusieurs décennies après l'arrêt de leur exploitation, d'imprégner les sols et l'environnement d'une pollution aux métaux lourds- arsenic, cadmium, cyanure. Ces dommages sur l'environnement affectent également les populations aux alentours du site pollué

prendre des centaines d'années. C'est notamment le cas des forêts vierges, nombreuses en Guyane, où les exploitations minières pourraient malheureusement se multiplier dans les décennies à venir. Aussi le présent Aussi le présent amendement vise-t-il à allonger la période de responsabilité des exploitants au regard des risques de l'après-mine, en tenant compte de la temporalité réelle de reconstitution des sols et des écosystèmes, notamment de la régénération du tissu végétal, qui s'étend sur des dizaines d'années.

L'article 20 du présent projet de loi permet donc l'extension, pour une durée de trente ans, des conditions d'exercice de la police résiduelle des mines après l'arrêt des travaux, afin de permettre à l'État de rechercher la responsabilité des exploitants en cas d'apparition de nouveaux désordres ou dommages. J'estime qu'il s'agit d'un bon équilibre. Je demande donc le retrait

Mme Raymonde Poncet Monge. L'exploitation minière industrielle et l'orpaillage illégal engendrent de nombreuses pollutions nocives pour la biodiversité et les populations, notamment en Guyane, au cours de l'exploitation, mais aussi de nombreuses années après

Cet amendement vise donc à doter l'État des moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'un plan de lutte efficace contre les pollutions minières, afin de prévenir les ruptures de digue, de faire face aux conséquences sanitaires, protéger les populations et de mener une évaluation publique des conséquences de l'activité minière, notamment en outre-mer. Quel

de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une stratégie unique, en articulant la répression avec des actions dans les domaines diplomatique, économique et social. J'ajoute que mon ministère finance l'augmentation de plus de 50

et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une définition de la mise en oeuvre d'une politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués.

par notre collègue a le mérite de clarifier la politique nationale de prévention et de gestion des sites et des sols pollués, en inscrivant les principes généraux de la protection des sols et des sous-sols au sein du code de l'environnement. Elle prévoit ainsi la prévention et la gestion des pollutions, y compris celles qui existent, et, surtout, la remise en état des sols dégradés, de manière à restituer à ces derniers un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts protégés par le code de l'environnement dans le cadre de la législation relative aux ICPE : la santé,

que l'évaluation du risque fondée sur les usages du site ; la connaissance des sources, vecteurs et cibles d'exposition, et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique. Mes chers collègues, les attentes de nos concitoyens sont fortes en la matière ; inscrire dans la loi ces principes généraux est un préalable indispensable.

Ces amendements visent à traduire la proposition n° 10 du rapport de la commission d'enquête du Sénat relative à la pollution des sols, qui a- je tiens à le souligner de nouveau -réalisé un travail considérable sur ce sujet.

l'amendement n° 960. La commission d'enquête dont nous avons parlé a souhaité mettre un terme aux asymétries existant entre le code minier et le code de l'environnement en matière de responsabilité des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux. notamment procédé à l'extension, aux exploitants de sites miniers, de l'obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ; à l'intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ; à l'extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante enfin, à l'intégration des travaux miniers dans l'autorisation environnementale, afin d'harmoniser les procédures administratives d'instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Notre constat a été, sans détour, celui d'une asymétrie entre le code de l'environnement et le code minier, en matière de responsabilité des exploitants. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de modifier le code minier, afin de soumettre les travaux de recherches et d'exploitation minières à un certain nombre d'obligations, dont le respect de la santé publique, ce qui convient à tout le monde- grande première -, et le respect des caractéristiques essentielles des sols. L'amendement vise surtout à harmoniser, pour la première fois, le régime de responsabilité des exploitants miniers, ce qui est une avancée importante. J'insiste sur ces éléments. Nous avons tous des expériences

1730. Je ne veux pas être redondant, l'objet est le même, il s'agit de mettre un terme aux asymétries existant entre le code minier et le code de l'environnement, en matière de responsabilité des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux, conformément à ce qui a été promu par notre commission d'enquête sénatoriale. Il s'agit, encore et toujours, de sécuriser la remise en état des sites et d'améliorer la surveillance des sols, car l'ambition, partagée par la quasi-unanimité des groupes politiques, est de mieux prévenir et de mieux gérer

Les intérêts halieutiques ont été également ajoutés dans ces intérêts protégés, à l'alinéa 9. Cet article permet désormais de rechercher la responsabilité des sociétés mères, grands-mères et arrière-grands-mères en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante. Le régime des garanties financières applicable à l'ouverture de travaux miniers a également été inscrit aux alinéas 11 à 23 de l'article 20. L'article 20 A, traité par la commission des affaires économiques et son rapporteur Daniel Gremillet, met en place un régime d'analyse environnementale, économique et sociale pour l'octroi, l'extension et la prolongation des permis de recherche et des concessions. L'article 20 , que nous examinerons ultérieurement, fait entrer les activités minières dans le champ de la responsabilité environnementale, défini par le code de l'environnement. Enfin, l'article 21, également traité par la commission des affaires économiques, habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin que, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers relève du régime de l'autorisation environnementale prévue dans le même code. Ces amendements identiques sont donc pleinement satisfaits. Je salue une nouvelle fois le travail réalisé par Mme Gisèle Jourda, l'ensemble des collègues de cette commission d'enquête et le président Lafon, car leurs recommandations ont inspiré certaines mesures proposées par le Gouvernement dans ce projet de loi.

se décharge sur les collectivités locales de ses responsabilités et surtout des dépenses y afférent, en ce qui concerne la surveillance et l'entretien des anciennes dépendances légales et, plus largement, des biens d'origine minière. Nous proposons donc la création d'un article relatif au transfert de biens, faisant expressément référence à l'article 72-2 de la Constitution. Cet amendement nous a été proposé par le collectif de défense des communes minières. Quel Les collectivités territoriales disposent d'un droit de priorité pour récupérer certaines installations hydrauliques de sécurité. Actuellement, le code minier prévoit que le transfert de ces installations est assorti du versement, par l'exploitant, d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative. Votre amendement vise à apporter une précision qui me semble intéressante au sein de l'article L. 163-11 du code minier, propos du transfert de biens d'origine minière de l'exploitant, de l'État ou de tout ayant droit à une collectivité locale. Il tend ainsi à sécuriser financièrement la reprise de ces biens par les collectivités,

de récupérer ces installations hydrauliques. Elles ont un droit de priorité, qu'elles peuvent utiliser si elles le souhaitent et en toute connaissance de cause, en sachant notamment le montant de la soulte qui leur sera versé pour solde de tout compte. Il est difficilement envisageable d'estimer une soulte qui correspondrait à un fonctionnement fonctionnement des installations, ainsi que les modalités de versement de cette soulte par l'exploitant. Si les collectivités ne souhaitent pas ce transfert, l'État reprendra ces installations. Le Gouvernement estime que la durée de dix ans fixée pour la soulte est proportionnée. Il n'y a donc pas lieu de compenser intégralement la reprise d'installations hydrauliques de sécurité

Actuellement, les pouvoirs publics sortent un grand parapluie administratif pour imposer leurs prescriptions Il en est ainsi d'une directive territoriale d'aménagement dans mon secteur minier, qui est bien connu : autour de la commune de Jarny, toutes les mines de fer ont été considérées de la même manière pour élaborer les prescriptions d'urbanisme. Pourtant, alors que,

Il vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme. Il est élaboré par l'État dans les conditions prévues par le code de l'environnement, sur le modèle du plan de prévention des risques naturels (PPRN), après une évaluation des aléas réalisée avec l'appui des établissements publics compétents. L'arrêté de prescription d'un PPRM ne contient pas, en lui-même, de disposition opposable créant des interdictions de construction. Une fois l'étude des enjeux et le projet de règlement réalisés, des concertations sont menées, puis une enquête publique précède l'approbation du PPRM, par arrêté préfectoral, qui peut être contesté par un recours contentieux. Dans le cas où le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines prescriptions d'un projet de PPRM et qu'il prend un arrêté d'application anticipé, il peut également y avoir un recours distinct pour excès de pouvoir.

Je suis désolé de devoir apporter à nouveau une précision. J'ai indiqué, en défense de mon amendement, qu'il existait une possibilité de recours lorsque la décision préfectorale d'approbation définitive du plan de prévention était rendue, mais cela peut prendre des années.

a abordé le volet du projet de loi relatif à la réforme du code minier. Il s'agit d'une réforme attendue depuis dix ans, qui fait consensus parmi les professionnels et les associations de protection de l'environnement. En effet, l'avant-projet de réforme a reçu l'accord unanime du Conseil national de la transition écologique.

enjeux de cette réforme sont multiples ; il faut, tout d'abord, actualiser un droit obsolète ; il faut aussi intégrer les enjeux environnementaux ; il faut enfin nous préparer à une concurrence mondiale pour l'accès aux ressources. Sur la méthode, cette réforme devait intervenir une très longue habilitation à légiférer par ordonnance. La commission a souhaité infléchir cette méthode en limitant l'habilitation dans le temps, en spécifiant les parties prenantes associées et en prévoyant une présentation devant le Parlement. Surtout, la commission a supprimé ou encadré quinze habilitations qui sont satisfaites par son propre texte ou par le Plus encore, la commission a inscrit directement dans la loi cinq dispositions issues de l'avant-projet de réforme : le caractère d'intérêt général des ressources, le principe de proportionnalité des procédures, celui de l'information préalable des collectivités, le registre électronique des titres et la recodification des reconversions. Elle a aussi conforté la sécurité juridique de certaines dispositions, à commencer par le contentieux minier, l'analyse environnementale et la lutte contre l'orpaillage illégal. Enfin, elle a posé le débat de la réforme de la fiscalité minière, qui est mal répartie entre les communes et conçue par rapport au cours des matières premières, comme celui de l'or, sujet que nous venons largement d'évoquer. Je souhaite que ce volet, tout à la fois infléchi et enrichi, aboutisse, car il y va de notre souveraineté minière.

à donner de la lisibilité aux opérateurs miniers, à conforter la concertation en amont des projets et à consolider la réforme du code minier. Il vise plus précisément à réformer la procédure de délivrance des permis exclusifs de recherche de gîtes contenant des substances de mines, en instaurant une phase de développement du projet avant la demande d'exploitation, afin de renforcer la concertation avec le territoire. Il tend aussi à instaurer une concertation du public pendant la phase d'instruction du permis exclusif de recherches et à adapter la durée du titre, désormais fixée à dix ans, à l'introduction des deux mesures précitées, ainsi qu'au processus d'évaluation environnementale, économique et sociale, prévu à l'article 20 .

issus de l'avant-projet de réforme, qui portent sur le caractère proportionné des procédures et sur l'information préalable des collectivités territoriales. D'autre part, le Gouvernement introduit des dispositions très substantielles, qui ne sont pas inutiles sur le fond, mais qui n'ont pas été soumises dans leur forme consolidée à l'avis du Conseil national de la transition écologique, une concertation conduite par la Commission nationale du débat public et des phases de développement des projets de géothermie ou de stockage. Surtout, il n'est pas de bon usage, madame la ministre, de soumettre des évolutions aussi importantes à la représentation nationale sans aucun échange préalable, alors que les auditions de la commission sur ce sujet ont débuté au début du donc émis un avis défavorable objet de garantir une plus grande sécurité juridique des dossiers. Il tend, à ce titre, à distinguer deux situations qui concernent deux étapes différentes du projet minier : l'ouverture des travaux miniers

Il vise à insérer deux alinéas ainsi rédigés : « L'analyse environnementale, économique et sociale définit le périmètre du cautionnement mentionné à l'article L. 155-1 du code minier. « Elle identifie les propriétés devant bénéficier de la caution et précise le mode de calcul et le montant de celle-ci. J'attire votre attention, monsieur le rapporteur : le code minier actuel prévoit bien, dans son article L. 155-1, des garanties financières sous forme de cautions, que l'exploitant doit, avant d'engager son exploitation sous des maisons ou des lieux d'habitation,

de l'analyse environnementale, économique et sociale. Cela permettrait d'informer et de rassurer les propriétaires d'habitation située au-dessus de la future exploitation minière, sur leur droit de bénéficier d'une garantie financière

au travail du rapporteur Pascal Martin, avec l'appui de la commission des affaires économiques. D'autre part, l'analyse environnementale, économique et sociale prévue dans le présent article précédera tout octroi, prolongation ou renouvellement de permis de recherche ou de concession. La commission demande donc le retrait de cet amendement

Il possède donc une expérience précieuse pour garantir une analyse et un accompagnement éclairé des dossiers. Compte tenu de cela et de la spécificité du territoire français en Guyane, nous pensons que l'ONF apportera un éclairage pertinent à l'octroi de titres miniers.

la suppression de l'avis conforme actuellement émis par l'ONF en Guyane sur les autorisations d'exploitation n'est prévue par aucune des dispositions relatives au code minier qui sont examinées dans le

pour avis. Sur l'initiative de la commission des affaires économiques, deux principes ont été inscrits « en dur » dans le présent article : le caractère proportionné des modalités d'instruction, d'information, de consultation ou de participation, l'information préalable des collectivités territoriales du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire. Il s'agit d'une demande très forte des collectivités. Mon amendement vise à intégrer à ces dispositifs les groupements de collectivités territoriales,

à l'octroi de concessions sur le gisement qu'il a découvert, sans que l'autorité compétente puisse s'y opposer. Nous avions déjà formulé une proposition identique lors de l'examen, en 2017, du projet de loi mettant fin à

la protection d'un environnement équilibré et respectueux de la santé, constitutionnellement garantie. Toutefois, dans l'hypothèse où le gisement découvert peut être exploité dans le respect des intérêts mentionnés à l'article précité, le titulaire du permis exclusif de recherche doit être le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d'exploitation. La nouvelle rédaction de l'article L 132-6 du code minier dérive d'un article du projet de loi portant réforme du code minier et portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit minier, sur lequel le Conseil national de la transition écologique a émis un avis favorable. Le sous-amendement

Monsieur le sénateur, la disposition que vous proposez correspond à l'approche que nous entendions défendre dans notre ordonnance, à savoir que le titulaire d'un permis exclusif de recherche est le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession sur le périmètre du permis exclusif de recherche qui lui a été accordé. Toutefois, il est nécessaire de déplacer ce nouveau dispositif dans la partie du code relative aux concessions, mieux adaptée, c'est-à-dire à l'article L. 132-6 du code minier. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour les permis exclusifs de recherche déjà accordés.

dans le cadre du droit commun. Par ailleurs, le projet de loi prévoit tout à la fois la modernisation du contentieux minier et l'association des collectivités territoriales à tous les stades de la procédure. Pour ce qui concerne l'amendement n° 1677 rectifié , le champ de l'article L. 142-4 du code de l'environnement, qui précise que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de préjudice direct ou indirect, n'est pas limité audit code. Il n'y a donc

zones sont parfois devenues inondables du fait d'un affaissement minier. Or le risque y reste considéré par les services de l'État comme un risque naturel. Pourtant, sans les travaux miniers, la zone ne serait pas inondable : ces derniers sont la cause déterminante du dommage. Aussi, une définition précise du dommage minier permettra de clarifier les responsabilités liées à l'exploitation minière. Pour que l'État cesse de jouer la montre avec les victimes de préjudices miniers, il convient aujourd'hui de clarifier la loi. Quel est l'avis de la

La commission des affaires économiques a, de surcroît, institué deux garde-fous protégeant les collectivités ou les citoyens concernés : d'une part, elle a introduit dans l'habilitation à légiférer par ordonnances l'exigence, pour l'État, de se porter garant de la réparation des dommages en cas de disparition ou de défaillance de l'industriel ; d'autre part, elle a prévu que chacune des ordonnances, dont celle sur le dommage minier, associe les parties prenantes, à commencer par les élus locaux.

les Maohis en Polynésie française, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie et, en Guyane, les Wayanas, les Lokono, les Tekos, les Kali'nas, ne me risquerai pas à prononcer le nom. Malheureusement, ces peuples et populations autochtones sont parfois les premières victimes des projets industriels qui s'imposent sur leur territoire, ainsi que de l'orpaillage illégal. Les modifications des écosystèmes engendrées par l'exploitation minière peuvent avoir des conséquences graves pour le maintien de leur mode de vie. Or la déstabilisation des structures sociales autochtones, à travers la destruction de leur espace de vie, aboutit souvent à l'effondrement de ces peuples, qui ne peuvent plus survivre. Il faut donc les protéger. D'ailleurs, leurs droits fondamentaux sont garantis par le droit international, qui dispose que les projets touchant les territoires des peuples et populations autochtones doivent recueillir préalablement

afin que le consentement libre, informé et préalable des populations et peuples autochtones soit pris en compte avant la délivrance de tout titre minier.

L. 161-1 du code minier, qui est modifié par l'article 20 du présent projet de loi, prévoit notamment que les travaux de recherches ou d'exploitation minières respectent les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou maritime et, plus généralement, à la protection des espaces naturels et des paysages de la faune et de la flore. Il renvoie également au code de l'environnement. Par ailleurs, les procédures préalables à l'exploitation minière permettent d'assurer un équilibre entre l'information des populations, la protection de l'environnement et le développement économique, notamment avec la procédure d'enquête publique et les concertations préalables. Enfin, je l'évoquais à l'instant, les commissions de suivi de sites permettront de garantir une bonne association du public

Nous regrettons ce choix d'autant plus que, si nous partageons l'objectif global de simplification, nous constatons également que son application est très variable selon les sujets. Il est donc fâcheux que cet argument ait été mis en avant à l'Assemblée Le présent amendement vise à revenir sur cette décision. Le conseil devrait être consulté sur l'élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol, l'ensemble des actes de nature réglementaire intéressant le secteur minier, les mesures de prévention liées aux risques miniers et le recyclage des métaux.

des « gueules noires », ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont donné leur vie pour la prospérité nationale, ceux-là mêmes qui ont été réprimés en 1948 après avoir- faut-il le rappeler ?

pour tous les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de l'Est, qui se retrouvent seuls face à un État qui joue la montre pour ne pas indemniser ces biens, ces vies fissurées par l'impunité des anciens exploitants. à l'article 20 , le conseil des mines, tel qu'il avait été proposé par la commission spéciale chargée de cette partie du texte. Il est indispensable d'entendre la voix des parties prenantes sur les questions minières passées et à venir.

relative à un tel titre a été déclarée recevable, afin de garantir l'information et une association large des publics concernés par l'exploitation minière. Ces commissions associent des représentants de l'État, des élus et des riverains, ainsi que les exploitants et les salariés des installations.

de la communauté scientifique. Ces deux ajouts permettent de satisfaire l'objectif, que je partage, d'une politique minière définie et pilotée en concertation avec les acteurs principalement concernés.

Ces infractions consistant majoritairement en l'activité d'orpaillage illégal, cette approche nous paraît trop restrictive : de nombreuses autres infractions mentionnées à la suite du code minier pourraient également être constatées par les agents de l'ONF,

l'étendue des forêts concernées en Guyane et de l'expertise de l'ONF, eu égard à la gestion et au maintien de ces forêts. C'est pourquoi nous proposons que l'ONF puisse constater l'ensemble des infractions prévues dans le code minier, et non seulement celles

Je rappelle que le dispositif initial ne comprenait aucune référence à quelque infraction que ce soit. Les infractions mentionnées correspondent à celles qui figurent dans tous les autres articles du projet de loi relatifs à la lutte contre l'orpaillage illégal.